Cette filière s’appuie sur un modèle unique au monde, ses ressources dépendant intégralement des paris hippiques, selon un monopole inchangé depuis 1891. Ces recettes font vivre les 40 000 personnes de la filière : professionnels agricoles, éleveurs, entraîneurs, C’est grâce à elles que peuvent être organisées 18 000 courses par an dans les 233 hippodromes répartis dans tous nos territoires. Pourtant, ce secteur vital fait face à une crise sans précédent. En dix ans, le PMU a perdu un tiers de ses clients.

Je propose le développement de nouvelles offres de jeux hippiques, dans le cadre de la fiscalité existante, tels que le et les paris sur des courses passées, mais anonymisées.

le sport populaire, nous proposons de relever à 20 % le taux de prélèvement sur les paris sportifs en ligne, à 16 % celui sur les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution, et à 12 % celui

Cet amendement s’inscrit dans une stratégie globale de réduction des risques. En effet, 40 % du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu

il y a quelques semaines. Les projets sélectionnés sont emblématiques et contribuent à la conservation d’un patrimoine naturel. À l’échelle locale, ils incitent les acteurs locaux à se saisir de la question écologique. Je pense en particulier au financement d’opérations pour le gypaète barbu, la tortue d’Hermann et les tortues marines en Martinique.

en matière d’emplois. Plusieurs dizaines de milliers de licenciements ont été enregistrés dans le monde ces deux dernières années. Dans ce contexte mondial, l’écosystème français n’est pas à l’abri. Des suppressions de postes ont également été annoncées sur notre territoire, même si la France continue d’occuper une place importante dans cette industrie très concurrentielle.

de cette industrie. Ce dispositif permet aux entreprises de création de jeux vidéo de déduire de leurs impôts une part des dépenses de production d’un jeu. Réformé en 2017, le CIJV montre toute son efficacité pour l’industrie française et internationale

les éditeurs de services de vidéo à la demande réalisant moins de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires. Cette mesure permettrait de conforter l’activité des petites plateformes françaises. Elle ne concernerait que les acteurs du marché de la vidéo à la demande les plus fragiles,

Pour les jeunes réalisateurs, il s’agit d’un passage obligé. Un certain nombre de dispositifs existent aujourd’hui pour financer ces premières réalisations et permettre l’émergence de nouveaux talents. C’est par exemple le cas d’aides versées par le CNC et les régions après de longues procédures. Ces procédures d’attribution, qui reposent sur des sélections faites par des comités de professionnels, favorisent le financement de projets d’auteurs déjà identifiés par le milieu, et donc la concentration des moyens sur quelques uns

Le crédit d’impôt visé permet à une société de production de déduire de son impôt sur les sociétés 25 % de certaines dépenses de production. À ce jour, les plafonds auxquels les œuvres concernées par ce dispositif sont soumises diffèrent selon leur nature. Ainsi, le crédit d’impôt au titre d’une œuvre audiovisuelle de fiction ne peut excéder 10 000 euros par minute produite et livrée si son coût de production est supérieur ou égal à 40 000 euros ; s’il s’agit d’une œuvre audiovisuelle d’animation, le plafond est alors fixé non pas à 10 000 euros, mais à 3 000 euros par minute. Ce plafond pour l’animation a été fixé dans la perspective d’une production destinée aux enfants et dont le préfinancement était principalement le fait d’acteurs français et européens.

Marco. En 2024, le Parlement s’est enfin saisi de la question des violences sexuelles et sexistes dans le milieu du cinéma : au Sénat, d’abord, avec l’adoption, en février dernier, de mon amendement visant à conditionner les aides du CNC à l’Assemblée nationale, ensuite, avec la création d’une commission d’enquête sur la question. J’ai déjà eu l’occasion de dire à quel point ce sujet est important, puisque le cinéma est un puissant lieu de représentation, qui participe à la diffusion de stéréotypes de genre. Cela tient aussi à la théorie du regard masculin : le fait que, des décennies durant, les films pour grand public ont été écrits par des hommes a eu un effet sur la manière dont les rapports entre hommes et femmes y ont été représentés. de l’affaire Weinstein aux États Unis, on sait également que cette domination masculine se doublait d’abus commis par des hommes en situation de pouvoir sur des femmes ou sur d’autres hommes moins puissants. cet amendement vise à conditionner le bénéfice du crédit d’impôt pour le cinéma au respect, par les sociétés de production, de dispositifs destinés à lutter contre les violences sexistes et sexuelles.

Cette taxe visait principalement les revenus tirés de supports physiques, comme les DVD et les salles de cinéma, mais elle a été rendue obsolète par les nouveaux modèles économiques du secteur et la montée en puissance des plateformes numériques. En 2021, la délégation aux droits des femmes du Sénat dressait un constat alarmant : en France, deux tiers des enfants de moins de 15 ans et un tiers des enfants de moins de 12 ans ont déjà eu accès à des images pornographiques.

Cet amendement vise à créer un « bon pour l’indépendance des médias » sous la forme d’un crédit d’impôt. En 2024, les États généraux de l’information ont réitéré le constat de l’inadaptation des aides à la presse versées par le ministre de la culture, ces aides étant en réalité concentrées sur les plus grands groupes de presse. À l’inverse, plusieurs médias indépendants ont cherché à garantir leur indépendance totale en n’en sollicitant pas Après l’ère des fausses nouvelles, nous entrons dans une ère de grande falsification des images et des récits, au moyen de l’intelligence artificielle. L’existence de sources d’information fiables et vérifiées est vitale pour le bon fonctionnement démocratique. Il importe donc de trouver des moyens de financer les médias indépendants sans transformer des aides en moyens de pression sur les rédactions. Il importe aussi d’encourager les citoyens à investir dans leur mode d’information et de leur faire prendre conscience qu’une information de qualité a un coût. C’est pourquoi l’économiste Julia Cagé proposait la création de bons pour l’indépendance des médias. De ce point de vue, le crédit d’impôt est idéal, car il permet une petite subvention publique sur l’initiative de chaque citoyen sans courir le risque d’immixtions politiques dans la définition de la ligne éditoriale.

cet amendement. Les revenus des artistes auteurs sont très irréguliers et leur permettent parfois de vivre pendant plusieurs années, en l’absence d’intermittences, dont ils sont exclus. C’est par exemple le cas des droits d’auteur versés à un scénariste ou des droits versés à un artiste plasticien après la vente d’œuvres à l’occasion d’une foire ou d’une exposition. C’est pourquoi le rapport de Bruno Racine, publié en 2020 et consacré à l’art et à la création, recommandait la mise en place de dispositifs de lissage fiscal des revenus, sur le modèle du dispositif existant pour les agriculteurs. Cet amendement d’appel

Monique de Marco. Cet amendement vise à traduire une proposition de notre collègue Sylvie Robert adoptée par le Sénat en 2023 et à permettre aux sociétés publiques locales de bénéficier des avantages fiscaux de soutien au mécénat d’entreprise prévus à l’article 238 du code général des impôts.

est probablement sous évaluée en raison d’une limite méthodologique qui ne permet pas de rendre compte du coût réel du mécénat pour l’État. Initialement prévu pour aider les artistes, l’art ou la culture, ou la culture, ce dispositif est désormais plutôt utilisé comme un outil d’optimisation fiscale. Avantageuses pour les entreprises, coûteuses pour le budget de l’État, ces dépenses fiscales représentent une perte de recettes et ne sont pas soumises à une évaluation de leur efficience ni à des objectifs de contrôle. Les gains que cet amendement permettrait de réaliser s’il était adopté pourraient être d’ailleurs directement réengagés au service du ministère de la culture, pour véritablement faire vivre notre démocratie culturelle.

et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé » de « déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition La déduction spéciale concerne les entreprises soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, ainsi que celles qui relèvent du régime des sociétés de personnes. Le présent dispositif contribue à faire entrer l’art dans l’entreprise. Il a largement été intégré, depuis quelques années, dans les démarches globales de responsabilité favorisant ainsi la diffusion et/ou la production d’œuvres, et contribuant à la sensibilisation des publics tant externes qu’internes, notamment par l’implication du personnel. En outre, si la constitution de collections d’œuvres d’art par les entreprises leur offre la possibilité de mettre en place un vecteur de communication externe, elle représente également un engagement sociétal et une amélioration du cadre de vie des salariés. De plus, la constitution d’une collection par les entreprises peut les conduire à entreprendre des actions de soutien aux artistes sous la forme de rencontres ou de résidences. Enfin, les entreprises détentrices de collection contribuent à la vitalité artistique par les dépôts qu’elles effectuent auprès des musées. Quel est l’avis de la commission ?

la réduction d’impôt sur le revenu accordée à tout particulier lorsque celui ci investit dans une entreprise de presse. L’objectif est de continuer à inciter le citoyen à participer au financement de la presse d’information politique et générale, tout en permettant aux entreprises de presse de diversifier leurs sources de capitaux. Pour les éditeurs, le développement de l’actionnariat salarié a réellement favorisé l’élargissement du vivier de donateurs. La fin de cette réduction d’impôt limiterait donc beaucoup les possibilités de levées de fonds complémentaires. Plus encore, la disparition de ce dispositif serait en contradiction avec les états généraux de l’information, qui ont placé au cœur de leur réflexion la question de la confiance entre les citoyens et les médias. La presse va mal

de participer au financement du renouvellement et de la diversité de la création éditoriale. La concentration du marché du livre d’occasion sur quelques plateformes – Amazon, Momox, Rakuten, eBay – se fait au détriment de la revente entre particuliers et du réseau des bouquinistes, en voie de disparition. Face à cette situation, la mesure redistributive que tend à proposer cet amendement vise à assurer la pérennité et l’équilibre de la filière du livre. ci repose en effet sur sa capacité à réinvestir une partie de la valeur créée dans le financement de la création artistique. Il s’agit de préserver notre modèle culturel, qui se caractérise par une production éditoriale abondante et diversifiée.

M. Adel Ziane. Cet amendement a pour objet d’exonérer les conjoints étrangers de Français de toute taxe liée à la délivrance ou au renouvellement de leur titre de séjour. Il s’agit de concrétiser une recommandation que le Défenseur des droits a formulée en 2014 et réitérée en 2016. en 2016. Contrairement aux conjoints étrangers de ressortissants européens résidant en France, les conjoints étrangers de Français doivent s’acquitter d’une taxe au moment de la délivrance et du renouvellement de leur carte de séjour. Le Défenseur des droits considère, à juste titre,

cache mal le désengagement financier notable de l’État. Le PLF pour 2025 prévoit d’aller encore plus loin. Le président du Comité des finances locales a bien souligné que la baisse cumulée des ressources des collectivités locales s’élèvera à près de 10 milliards d’euros. Cette situation n’est pas tenable. Les collectivités locales sont les garantes des services publics. Ce sont elles qui assurent au quotidien, vous le savez tous, la proximité nécessaire pour maintenir le lien social et pour répondre aux attentes concrètes des habitants. À rebours des accusations sur leur supposée mauvaise gestion, elles ont apporté une contribution majeure au redressement des finances publiques. Nous demandons une augmentation significative de la dotation globale de fonctionnement. Ce concours financier est non pas un luxe, mais une nécessité. Loin de représenter une charge pour l’État, les collectivités locales sont une richesse. Chaque euro qu’elles investissent produit de l’activité économique, crée de l’emploi et améliore la qualité de vie.

l’an dernier, elle passe à 487 millions cette année. Alors que les gels de dotation entre 2018 et 2022 se sont traduits par une pénalisation financière

On pérennise ainsi les deux hausses successives de 320 millions d’euros en 2023 et en 2024, qui ont fait suite à treize années de baisse. Je rappelle que 82 % des communes ont connu une stabilité et une progression de leur DGF en 2024 par rapport à 2023, ce qui n’était pas le cas au cours des mandatures précédentes. On avait notamment assisté à une importante

de bonne gestion quand on dresse le bilan des nombreuses décisions unilatérales prises par l’État depuis quelques années pour accroître les

et 2024, il renoue ainsi avec le gel appliqué de 2018 à 2022. Le présent amendement tend, au contraire, à revaloriser la DGF du bloc communal à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation pour 2025, soit une hausse de 1,8 %. La DGF des communes et des EPCI augmenterait ainsi d’environ 341 millions d’euros par rapport à 2024.

qui ne disposent plus de dotation forfaitaire. La solution technique consistant à faire participer les communes sans dotation forfaitaire au financement des dotations de péréquation directement par prélèvement sur leurs douzièmes se révèle également inopérante, dans la mesure où l’article 64 du présent projet de loi prévoit par ailleurs qu’elles seront ponctionnées à hauteur de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement, un niveau plafond selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Afin d’éviter que le financement de la péréquation soit

monsieur le ministre, il faut réduire les déficits, mais pas sur le dos des collectivités. Je répète qu’elles ne sont pas responsables de la situation financière ! Les

l’inflation était égale à zéro. À l’époque, les collectivités avaient encore conservé une forme d’autonomie fiscale. Aujourd’hui, tout cela a disparu l’inflation est beaucoup plus élevée et l’autonomie fiscale et financière, à la suite de vos décisions, a été quasiment réduite à néant. Les marges de manœuvre des élus locaux se sont donc forcément considérablement réduites. Par ailleurs, il faut insister sur l’effet de ciseaux

stabiliser la DGF ne signifie pas qu’il n’y aura pas de contribution financière des collectivités territoriales par ailleurs ! Ne faites pas semblant de ne pas comprendre, vous le savez très bien.

Une augmentation aussi brutale met en péril la soutenabilité budgétaire des collectivités, déjà affaiblies par un contexte financier marqué par la non indexation de la DGF sur l’inflation. Par ailleurs, ce mécanisme se révèle incohérent dans sa mise en œuvre coopération intercommunale (EPCI) les plus intégrés, dont l’effort de mutualisation est pourtant reconnu par une dotation d’intercommunalité majorée. Cette contradiction, monsieur le ministre, illustre une répartition financière mal pensée, qui va à l’encontre de l’équité dont vous vous réclamez. Enfin, cette ponction discrédite fortement la parole de l’État,

Espagnac, pour présenter l’amendement n° I 149. En 2024, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions représente 467 millions d’euros et constitue une ressource à part entière de leur budget.

région a été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé, en 2021 et 2022, le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli », « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de 5,9 % en 2023, ce qui représente une diminution de 400 millions d’euros, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1

prévu par le PLF pour 2025 porte à 38 % la baisse de la DCRTP des régions. Cet effort apparaît disproportionné au regard de leur situation financière. Afin de préserver les ressources à la formation professionnelle, au fonctionnement des lycées, aux aides aux entreprises et à la capacité d’investissement des régions, dans un contexte de fort ralentissement de leurs recettes, le présent amendement vise à figer le montant de la DCRTP sur celui qui a été versé aux régions en 2024. La parole est à Mme Brigitte Devésa,

à 467 millions d’euros. Évidemment, pour 2025, une nouvelle baisse est prévue, d’un montant de 189 millions d’euros, ce qui équivaut à 40 % des recettes de cette taxe. Or les régions, comme les départements, sont déjà en difficulté financière. En effet, la Cour des comptes a constaté, pour celles ci, une situation financière en repli, qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement. Les régions ont vu leur épargne brute baisser

6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui qui a été constaté lors de la crise sanitaire. Dans ce contexte, le présent amendement vise à figer le montant de la DCRTP sur celui qui a été versé aux régions en 2024, afin de préserver les ressources de ces collectivités.

à leur niveau de 2024.

J’insiste sur le fait que cette dernière dotation, instaurée lors de la suppression de la taxe professionnelle, visait précisément à compenser, de manière intégrale et pérenne, les baisses de recettes des collectivités les plus perdantes dans cette réforme. Pour le bloc communal, il s’agissait principalement de communes et d’EPCI situées sur des territoires industriels ou fragiles. Quant aux fonds de péréquation, ils sont versés à des communes et EPCI défavorisés au regard des critères de ressources et de charges. Ainsi, ils ont une visée de péréquation au sein des départements éligibles.

Le scrutin est ouvert.

du RSA. Je propose donc d’abonder de 463 millions d’euros le fonds de sauvegarde des départements, créé par la loi de finances pour 2020 et déjà mobilisé en 2024 à hauteur de 100 millions d’euros. Sa dotation actuelle ne serait estimée qu’à 37 millions d’euros, ce qui est largement insuffisant pour apporter une garantie de solvabilité à la quinzaine de nouveaux départements qui devraient être déclarés en difficulté cette année. Le montant de 463 millions d’euros qui vous est proposé a été estimé sur la base de calculs réalisés pour déterminer les moyens nécessaires au rétablissement de la situation financière des départements les plus vulnérables. L’amendement

même si, à terme, il conviendrait de repenser le financement de cette collectivité singulière et indispensable à la République.

élargissement de la prime à tous les personnels du secteur sanitaire, social et médico social privé à but non lucratif doit rester un objectif de justice sociale, indépendamment de la réalité financière des collectivités chargées de son versement.

J’attire votre attention sur un sujet capital pour la Corse, et je pèse mes mots : la dotation de continuité territoriale (DCT). Comme vous le savez, chaque année, les élus corses demandent au Gouvernement d’abonder cette enveloppe, gelée depuis 2009.

Pour l’année 2024, la perte de recettes est alarmante : elle atteint les 53 millions d’euros. En 2023, la TVA n’a représenté que 20 % des recettes de fonctionnement de la collectivité de Corse, contre 55 % dans les régions métropolitaines. Cette exclusion de la DCT des ressources transformées en fraction de TVA a créé un déséquilibre structurel, laissant la collectivité de Corse avec des recettes bien inférieures à celles de ses homologues continentaux. Cette situation est intenable et limite notre capacité à financer les services publics essentiels, exacerbant ainsi les difficultés de nos concitoyens et nos acteurs économiques.

un ajustement automatique face à l’inflation et aux besoins croissants de nos services publics. Enfin, nous pourrions ainsi en finir avec la rupture d’égalité qui découle de ce gel.

primordial pour la Corse. En effet, si un avion ne décolle pas, sachez, mes chers collègues, que ce sont des centaines de personnes qui devaient se faire soigner qui restent coulées au sol. Si un bateau n’arrive pas

et une restriction du périmètre des dépenses éligibles, soulève des préoccupations majeures tant dans son principe que du point de vue de la réalité de terrain. Rappelons d’abord que le FCTVA n’est pas une subvention, mais une juste compensation de la TVA supportée par les collectivités dans le cadre de leurs investissements. Réduire le taux forfaitaire de remboursement de 16,40 % à 14,85 % revient à faire peser une charge supplémentaire de 800 millions d’euros par an sur nos collectivités, qui sont déjà fragilisées par des contraintes budgétaires croissantes. En outre, l’exclusion de certaines dépenses du périmètre éligible – entretien des bâtiments publics, voiries, réseaux ou encore prestations informatiques – est tout aussi préoccupante. Ces dépenses, bien qu’elles ne relèvent pas strictement de l’investissement, sont essentielles à la continuité des services publics et à la modernisation des infrastructures locales. Les collectivités investissent non pas pour elles mêmes, mais pour répondre aux besoins de leurs habitants. Au delà de ces considérations techniques, cette réforme envoie un signal négatif dans une période de crise économique où chaque euro d’investissement local compte pour relancer l’activité et maintenir l’emploi.

Cet article modifie, pour 2025, le taux remboursé aux collectivités territoriales au titre du FCTVA, pour une moindre compensation estimée à 800 millions d’euros.

Cette mesure, si elle était adoptée, constituerait incontestablement un signal négatif pour les investissements des collectivités locales, lesquels représentent tout de même plus de 70 % de la commande publique. Un tel dispositif n’est pas acceptable.

dans les collectivités d’outre mer. Par ailleurs, la complexité des opérations d’aménagement inhérente à la quête de la réalisation de l’objectif du zéro artificialisation nette exige des financements durables et suffisamment dotés pour assurer l’équilibre de l’équation nécessaire à la diminution de l’empire foncière. Quel est l’avis du Gouvernement ?

sur l’article. L’article 31 entérine une atteinte majeure à l’autonomie financière des collectivités territoriales. Après avoir vu des pans entiers de leur fiscalité supprimés ces dernières années, qu’il s’agisse de la taxe d’habitation ou de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, doivent désormais faire face à la remise en question de la compensation de la TVA. Cette réforme, qui stabilise en valeur les fractions de TVA affectées aux collectivités pour 2025, se traduira par une perte nette estimée à 1,1 milliard ou 1,2 milliard d’euros.

Depuis plusieurs années, les collectivités locales sont devenues de plus en plus dépendantes de la TVA, un impôt d’État, en raison des réformes successives. Cependant, cette dépendance à un impôt national représente un risque majeur : elle fragilise l’autonomie financière des collectivités. En effet, contrairement aux impôts locaux comme la taxe d’habitation ou la CVAE, dont les collectivités avaient la maîtrise, la TVA est soumise à des ajustements unilatéralement décidés par l’État. Cette réforme, en imposant les transferts, en est la preuve éclatante.

Au delà des chiffres, cet article est aussi un signal politique inquiétant. Renoncer à compenser pleinement les pertes de fiscalité des collectivités, c’est miner la confiance entre l’État et les territoires, c’est affaiblir l’autonomie de décision des élus locaux, c’est limiter leur capacité à répondre aux attentes de leurs concitoyens. Mes chers